notre pays a de nouveau été touché mardi soir par une lâche attaque terroriste. Un individu, qui reste recherché à cette heure, a semé la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg, une ville symbole. Le bilan humain est lourd : trois personnes sont décédées, une autre est dans un état très critique et treize sont blessées, dont plusieurs grièvement. Au nom du Sénat tout entier, je tiens à adresser nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nos pensées vont aux blessés et à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble de nos compatriotes strasbourgeois. Je veux dire notre solidarité à Roland Ries, notre ancien collègue, maire de Strasbourg, et à tous nos collègues du Bas-Rhin. Je tiens à saluer le professionnalisme des forces de sécurité, déjà mises à rude épreuve depuis 2015. Face au terrorisme, nous devons impérativement demeurer unis dans un esprit de responsabilité. Je vous invite à observer un instant de recueillement en hommage aux victimes de cette attaque.

je vous remercie pourriez-vous éclairer le Sénat sur l'organisation de l'ordre du jour à la suite des annonces faites par M. le Président de la République ? Quels sont les ajustements attendus d'ici à la suspension de nos travaux ?

capitale de Noël, des innocents sont encore tombés, des familles sont encore endeuillées. Et la liste des victimes du terrorisme dans notre pays continue de s'allonger.

Bien sûr, nous savions que la menace qui plane depuis maintenant des années sur notre pays n'avait pas disparu. Mais elle nous semblait peut-être moins palpable, moins oppressante au quotidien. Le drame de mardi nous nous rappelle violemment combien elle est toujours d'actualité. Je veux saluer le courage et l'engagement de nos forces de l'ordre et de sécurité, de nos services de renseignement. Leur travail acharné, souvent dans l'ombre, nous protège au quotidien. Mais il ne peut pas tout éviter. Je veux également saluer le dévouement et le professionnalisme de nos équipes médicales et d'urgence. Le criminel qui a sévi à Strasbourg était connu de la police et de la justice. Il était « fiché S » et inscrit au Ainsi, certains ne manqueront pas, une fois encore, de relancer de vaines polémiques sur le sort qu'il faudrait leur réserver ... Nous ne voulons pas aller sur ce terrain. En revanche, on doit s'interroger sur ce type de profils qui basculent de la délinquance de droit commun à la radicalisation, notamment lors de leurs passages en prison. Depuis plusieurs années, on nous a vendu la déradicalisation comme étant la solution pour enrayer le risque terroriste. Malgré les nombreuses tentatives en la matière, les résultats sont peu probants, voire nuls. Monsieur le Premier ministre, peut-on encore espérer quelque chose de ces méthodes ? Et, avec le souci de mieux protéger nos concitoyens, quelles solutions alternatives votre gouvernement propose-t-il ? La parole

terroriste endogène d'individus présents sur notre territoire et qui passent à l'acte. Vous avez raison de souligner que les services de renseignement, les services de police et de gendarmerie sont très concentrés pour lutter contre cette menace : ils la prennent très au sérieux et ne baissent jamais la garde. Comme vous le savez, il est essentiel de pouvoir détecter ces individus, de pouvoir les suivre au plus près. C'est à cette fin qu'est tenu un fichier de suivi des individus radicalisés ; c'est à cette fin que les objectifs sont répartis entre tous les services de renseignement, pilotés dans chaque département par les préfets, dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux. Ce travail est effectué au plus près, il a été renforcé par une augmentation des moyens humains et il va se poursuivre tout au long du quinquennat, puisque 1 900 emplois seront créés à cette fin.

et suivi par un service de renseignement de manière exhaustive, mais, malheureusement, jamais il n'est apparu de velléité de passage à l'acte. Je peux vous garantir que ce suivi a été fait sérieusement, et qu'il se poursuivra pour l'ensemble des objectifs. Christophe Castaner et moi-même le rappelons

de terrain pour prendre en compte les individus radicalisés les plus fragiles et mettre en place des actions de déradicalisation. Il y a une action répressive et une action préventive qui sont menées. Ces actions se poursuivront avec beaucoup de détermination.

au nom des sénateurs du groupe La République En Marche, je tiens à me joindre à la solidarité unanimement exprimée dans cet hémicycle à l'égard des victimes du terrible attentat survenu à Strasbourg. Je tiens également à remercier les pompiers et les forces de l'ordre pour le travail remarquable qu'ils réalisent quotidiennement en faveur de la protection et de la sécurité des Français, en particulier ces dernières semaines, à la suite des nombreuses manifestations qui ont émaillé notre territoire. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a décrété lundi « l'état d'urgence économique et sociale » après trois semaines de crise des « gilets jaunes » dans l'Hexagone et en outre-mer, notamment à l'île de la Réunion. Réunion. « Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail ; sur ce point, nous sommes allés trop lentement », a affirmé le Président de la République. Cette volonté affichée du chef de l'État se traduit par des annonces fortes et concrètes : l'annulation immédiate des taxes sur le carburant, une super-prime à la conversion, la défiscalisation des aides régionales et l'élargissement du chèque énergie. Ensuite, dès le début de l'année prochaine, un salarié au SMIC bénéficiera d'un gain mensuel de cent euros, les retraités percevant moins de 2 000 euros par mois seront exemptés de la hausse de la CSG et les heures supplémentaires déjà désocialisées dans le budget de 2019 seront défiscalisées. Enfin, la prime de fin d'année versée par les entreprises ne supportera ni impôts ni charges. Il s'agit là de mesures considérables et d'un effort budgétaire important pour la Nation. Les travailleurs et les retraités les plus modestes méritent toute notre attention. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de la prochaine mise en oeuvre de telles mesures. Toutefois, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser les modalités concrètes d'application de ces annonces ?

prises par le Gouvernement et annoncées par le Président de la République concernant la question du pouvoir d'achat et la question de la transition écologique. M. le Premier ministre a précisé

il faut préciser que la prime d'activité, qui a été évoquée comme l'un des moyens d'augmenter le revenu des salariés payés au niveau du SMIC, est accessible tant aux salariés du secteur privé qu'aux salariés du secteur public. Il faut préciser aussi que la défiscalisation des heures supplémentaires sera applicable aux salariés du secteur privé comme aux agents publics. En ce qui concerne la CSG, il s'agit d'exonérer de la hausse de l'année 2018 les retraités qui, pris individuellement, ont une retraite inférieure à 2 000 euros net par mois. Cela concerne 3,7 millions d'entre eux. La moitié des retraités qui ont vu leur CSG augmenter en 2018 verront donc cette augmentation annulée au cours de l'année 2019.

Monsieur le ministre, en cette période de tension sociale, la question du pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations de nos concitoyens. À notre sens, cela passe nécessairement par le fait de donner les moyens à chacun de vivre dignement de son métier. On doit le souhaiter aussi pour nos agriculteurs. C'est vrai ! Les États généraux de l'alimentation ont suscité de grands espoirs. La loi ÉGALIM est sortie de ces discussions avec pour principal objectif de rééquilibrer les relations commerciales et d'améliorer la rémunération des agriculteurs. Pour l'application de certaines de ses dispositions, nous attendons des ordonnances. La première, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions, a été présentée hier en conseil des ministres et publiée aujourd'hui au. C'est une bonne chose, car les mesures portées par cette ordonnance vont dans le sens d'un meilleur rééquilibrage des relations commerciales au profit des producteurs.

et se déroulent dans des conditions difficiles. Il faut vraiment accélérer la mise en oeuvre de ce texte. Dans l'intérêt de nos agriculteurs, nous sommes tous attachés à faire en sorte que cette loi atteigne ses objectifs.

travailler à l'augmentation de la rémunération des agriculteurs. Cela fait maintenant des années que les négociations commerciales se passent mal pour la profession agricole.

le Sénat, sur l'initiative du groupe Les Républicains, avait voté un amendement en faveur de l'augmentation des droits d'inscription universitaires pour les étudiants non communautaires. Vous vous y étiez opposée, madame la ministre. de la commission mixte paritaire, votre collègue Gabriel Attal avait repoussé la mesure en déclarant : « Les étudiants étrangers deviennent ensuite les ambassadeurs de la France dans leur pays et transmettent des valeurs. » Le Premier ministre a annoncé, le mois dernier, que le montant de ces frais serait multiplié par pour la licence. Pourquoi le Gouvernement a-t-il ainsi changé d'avis ? La procédure Parcoursup a fait subir aux bacheliers des filières technologiques et professionnelles de graves discriminations d'accès à l'enseignement supérieur. Notre groupe

de l'énergie avec laquelle vous portez un point de vue dont j'ai pu vous démontrer, notamment en commission, qu'il était totalement erroné. Parcoursup, c'est 23 % de bacheliers professionnels en plus dans les BTS,

En ce qui concerne les étudiants internationaux, là encore, que de simplifications ! Ce que le Premier ministre a annoncé, c'est un plan d'accueil des étudiants internationaux, intitulé « Bienvenue en France », qui a été coconstruit par trois ministères.

paieront un tiers du coût complet de leurs études et ceux qui paieront, c'est-à-dire ceux qui viendront dans des conditions particulières fixées par les établissements, contribueront au meilleur accueil de 100 % des étudiants. Incroyable

pour le Gouvernement. La communauté universitaire et les étudiants ne se satisferont pas de vos réponses techniques. Ils considèrent que l'annonce gouvernementale, sans aucune concertation, est un affront porté à la tradition universitaire française. Ils vous demandent maintenant de réaffirmer l'universalité de la pensée française, le rôle essentiel des universités pour en assurer la diffusion et, surtout, l'abandon immédiat de toutes les mesures discriminatoires d'accès à l'enseignement supérieur. La

socialiste et républicain. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'intérieur, quand les nuits s'allongent jusqu'au solstice d'hiver, quand les brouillards de décembre nous privent de soleil dans ces jours trop courts, les lumières et les décors de Noël nous libèrent de la déprime. Cette tradition des pays du Nord est forte en Alsace. Elle fut païenne, puis chrétienne et donne à tous un esprit de fête, de chaleur et de fraternité. Cette ambiance vient d'être brisée à Strasbourg en ce 11 décembre. Un jeune homme né à Strasbourg, issu des quartiers de la ville, a donné la mort et blessé grièvement des touristes et des habitants, y compris un Afghan membre d'une communauté musulmane. Mes premières pensées comme celles de tout le monde, et je vous remercie tous de votre solidarité, vont d'abord, bien entendu, aux innocentes victimes et à leurs proches, à ces vies brisées au coeur de la fête. Notre gratitude va aux forces de l'ordre, si fortement sollicitées durant ces semaines de troubles, et elles le seront encore. Notre gratitude va aussi aux services de secours et de soins. Notre espoir, monsieur le ministre, est que les forces de l'ordre arrivent à arrêter cet assassin, car, aujourd'hui, l'angoisse persiste au coeur de la ville. Je crois toutefois comprendre, à travers les informations que nous recevons sur nos smartphones, qu'une opération du RAID est en cours, ce qui serait une bonne nouvelle.

pour aider les services de renseignement à mieux distinguer les personnes présentant le plus de risque ? Dans d'autres pays européens, et notamment en Belgique, on est en train de revoir les systèmes, et en particulier les algorithmes ; c'est peut-être une piste. Je le dis sans vouloir polémiquer parce que notre intérêt à tous c'est que la sécurité puisse être renforcée.

Il faut les entendre, répondre à leur inquiétude et les soutenir. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que les agriculteurs qui ont subi des pertes très importantes à cause de la sécheresse seront indemnisés rapidement ?

les agriculteurs souffrent beaucoup et le Gouvernement sera au rendez-vous pour répondre à leur détresse. Plus largement, vous avez raison de dire que, en dehors des mesures sporadiques ou conjoncturelles liées aux aléas climatiques, sanitaires ou autres, il est important de regarder comment l'agriculture française

après Claude Kern et Jacques Bigot, permettez à un troisième sénateur alsacien, demeurant à Strasbourg, de s'exprimer après le drame qui a endeuillé sa ville. Au nom du groupe Les Républicains, je veux à mon tour m'incliner devant les victimes et dire notre compassion à l'égard de leurs familles et de leurs proches. Je veux également réaffirmer notre soutien et rendre hommage aux forces de l'ordre qui, injustement malmenées ces derniers temps, font un remarquable travail de protection de la population tout au long de l'année, particulièrement durant la période des fêtes de fin d'année. Strasbourg, capitale des droits de l'homme, capitale de l'Europe des valeurs, comme le dit son maire, a été touchée au coeur

Le symbole, mes chers collègues, est fort et la blessure est profonde. Pour autant, je veux affirmer solennellement que, malgré la barbarie qui les frappe, les Alsaciens ne renonceront pas à porter leurs valeurs d'humanisme, que d'aucuns voudraient voir disparaître.

de la répétition de cette chaîne mortifère, qui commence par de la délinquance de droit commun et se poursuit par de la récidive et de la multirécidive- vingt-sept fois ! -, puis par une radicalisation en prison, puis fichier S, et, enfin, trop souvent, la tentation du passage à l'acte terroriste. Les exemples sont nombreux, je ne veux pas les citer ici pour ne pas faire la promotion de leurs auteurs. Monsieur le Premier ministre, on sait que 450 détenus radicalisés seront libérés l'année prochaine.

a évoqué jeudi dernier dans cet hémicycle notre vision de la situation et nos propositions pour y répondre. Lundi dernier, le Président de la République a annoncé diverses mesures, elles sont essentiellement à destination que de nombreux autres Français souffrent et se sentent délaissés. Ils vivent également dans la précarité, avec de faibles ressources ; je pense à des artisans, agriculteurs, pêcheurs et professionnels indépendants qui connaissent aussi de graves difficultés et s'inquiètent pour leur avenir et celui de leur famille. Je pense encore aux projets de reprises d'Ascoval, dans le Nord, et de Ford à Blanquefort, pour lesquels le ministre de l'économie et des finances est particulièrement mobilisé. Nous aimerions connaître vos propositions pour ces Français, qui ressentent tout autant le ras-le-bol fiscal et social. Par ailleurs, le coût des mesures annoncées est élevé, au moins 10 milliards Éviter la forte dégradation des comptes publics est impératif. Au Sénat, nous appelons de longue date à une réduction de la dépense publique, mais aussi à une lutte accrue contre la fraude fiscale et à une taxation des entreprises qui optimisent ou masquent leurs profits. masquent leurs profits. Quelles mesures complémentaires le Gouvernement entend-il prendre pour que, outre les attentes liées au pouvoir d'achat, des réponses soient également apportées à ce sentiment d'injustice fiscale et sociale ?

pour tenir les comptes publics et pour nous rapprocher le plus possible des 3 % de déficit public- c'est notre engagement européen et nous y tenons. Nous ferons des propositions, dans les jours qui viennent, pour aller dans ce sens. Raison de plus pour lutter contre l'optimisation fiscale, raison de plus pour taxer les géants du numérique, raison de plus pour mettre en place un minimum d'imposition pour ces multinationales qui s'installent à l'étranger et ne payent pas leur juste imposition en France. Nous le ferons.

Je suis révolté, je suis écoeuré par cette décision, qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer la lâcheté de Ford, à qui je demande de parler depuis trois jours et qui n'a même pas eu le courage de prendre le ministre de l'économie et des finances au téléphone. Je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit, dans ce communiqué, que l'offre de reprise de Punch n'est pas crédible, alors que nous y travaillons depuis des mois avec les salariés et Punch. C'est une offre industrielle crédible, solide, qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort. Et je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site de Blanquefort. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage, parce qu'ils avaient accepté de réduire leurs salaires

! Je veux profiter de la représentation nationale pour appeler solennellement Ford à réviser sa décision et à accepter une reprise par Punch, qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort à Bordeaux.

Il est important que les promesses annoncées soient effectivement tenues. La parole est à M. Éric Gold, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. et Social Européen. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elle reprend pour partie une question qui a déjà été posée. Madame la ministre, le 10 décembre, alors que plusieurs facultés étaient bloquées et que des étudiants rejoignaient les manifestations lycéennes, la Conférence des présidents d'université a publié un communiqué, demandant au Gouvernement de suspendre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens et de mettre en place un groupe de travail sur le sujet. Ce communiqué fait suite à l'annonce, par le Premier ministre, du plan Bienvenue en France, qui vise à conforter l'attractivité de la France dans le domaine universitaire. Je m'associe pleinement à votre ambition d'accueillir plus d'étudiants étrangers pour demeurer au rang des premières nations en matière de mobilité étudiante. Toutefois, cet objectif peut sembler contradictoire avec l'augmentation subite des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, qui interviendra dès la rentrée 2019. Pour les étudiants de licence, c'est 2 600 euros de plus à débourser et pour les étudiants de master et de doctorat, environ 3 500 Si certains pourront faire face, d'autres devront nécessairement renoncer à leur projet. À l'Université Clermont-Auvergne, l'UCA, plus de 5 000 étudiants étrangers sont accueillis chaque année. Ils participent à la renommée et à l'excellence de ce site, ainsi qu'à celles de l'ensemble des universités françaises. Cette dynamique est par ailleurs une chance et représente beaucoup pour de nombreux territoires, qui s'inquiètent des conséquences possibles d'une telle mesure. Vous avez annoncé vouloir tripler le nombre de bourses, mais elles ne pourront pas permettre d'accueillir tous les étudiants modestes, Ce sont ainsi les intellectuels, les ingénieurs et les cadres de demain que nous laissons partir. Exactement ! Ils étaient déjà 80 000 Africains à étudier en Chine cette année, où ils bénéficient de la scolarisation et du logement gratuits, ainsi que d'une bourse mensuelle de 400 euros. Cette relation privilégiée avec un continent à la dynamique puissante, relation construite du fait de notre histoire et de notre langue, doit absolument être préservée malgré des impératifs économiques que nous comprenons bien.

Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Gold, le premier objectif de ce plan Bienvenue en France est de doubler le nombre d'étudiants internationaux

déjà présents sur le territoire, qui sont en train d'étudier et pour lesquels, bien sûr, les droits d'inscription ne sont pas modifiés, mais aussi ceux qui seront exonérés des nouveaux droits. De ce point de vue, j'ai rappelé à la Conférence des présidents d'université que seuls les conseils d'administration des universités avaient le pouvoir d'exonérer les étudiants internationaux. est très important de construire cette stratégie d'accueil et d'attractivité. C'est pourquoi nous avons aussi travaillé à la mise en place d'un label correspondant à cette qualité d'accueil, label pour lequel plus de soixante-dix établissements se sont déjà positionnés. Vous

exonérés des droits d'inscription des universités chinoises, qui s'échelonnent entre 1 800 et 4 500 euros par an. Notre politique est de tripler le nombre des bourses de façon à pouvoir accueillir les étudiants internationaux.

Les mouvements que nous connaissons depuis ces dernières semaines nous rappellent, si besoin était, à quel point les salariés de ce pays peuvent se sentir dépréciés quant à leurs conditions de travail et, surtout, de rémunération. Ils nous rappellent également que la transition énergétique ne peut se faire uniquement à coup de taxes, dont les plus modestes sont souvent des victimes. Mais ces mouvements en disent long également sur le niveau de défiance à l'égard de nos gouvernants. Ils reflètent ainsi le sentiment que ceux-ci ne s'intéressent pas au quotidien de leurs concitoyens. Par conséquent, tous les dossiers dont nous vous saisissons, mesdames, messieurs les ministres, doivent se voir apporter des réponses concrètes. Je vais prendre un exemple précis, celui de la situation Aujourd'hui, dans mon département, nous sommes à la veille d'une catastrophe économique. Plus de 30 millions de mètres cubes de bois restent sur pied, alors qu'ils devraient être mis sur le marché, rendant ainsi la ressource rare et donc beaucoup plus chère. Tous les maillons de la chaîne- scieries, usines de productions de papier et autres -sont ainsi affectés. Au bout de la chaîne se trouvent des ouvriers et des employés dont les salaires ne sont pas élevés et pour lesquels la forêt reste la seule richesse. le bois produit en France, celui que l'on n'importe pas, est avant tout un enjeu de transition énergétique et écologique. Nous sommes donc au coeur du sujet : l'adaptation de notre modèle économique aux impératifs environnementaux, le respect des entreprises et de leurs salariés, le maintien de l'emploi en zone rurale. Voilà, dans le contexte actuel, une étude de cas concrète, si j'ose dire ! Après la tempête Klaus, les propriétaires ont bénéficié d'aides publiques très importantes et continuent à en bénéficier par le biais d'exonérations au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Charge à eux de respecter des plans de gestion. Vous venez de signer, monsieur le ministre, un contrat de filière plein de promesses, concernant notamment la mobilisation de la ressource. Ma question est simple, monsieur le ministre : quand prendrez-vous les mesures nécessaires au respect de ces plans de gestion, c'est-à-dire tout simplement au respect de la loi ? Dans mon département, la forêt engendre 4 000 emplois directs.

par l'ensemble des signataires. Je devais me rendre aujourd'hui à l'assemblée générale de la fédération nationale du bois, mais j'ai souhaité être présent ici même pour répondre à votre question. Oui, le contrat de filière a été signé, oui, nous nous engageons, des mesures ont déjà été prises.

Ignorant les avertissements de notre assemblée, vous vous êtes opposés à ces propositions. L'an dernier, nous avions signalé les difficultés rencontrées par les retraités les plus modestes à la suite de la hausse de la CSG, que nous avions contestée. Cette année, nous avons, dans le PLFSS, refusé la désindexation des pensions de retraite, que vous avez pourtant confirmée. L'an dernier, comme cette année, dans le cadre de l'examen du budget, nous avons pris des mesures de lutte contre la fraude à la TVA, ainsi que des mesures de lutte contre la fraude aux dividendes, et le Gouvernement n'a pas donné son accord.

Depuis quelques jours, les choses ont changé. Depuis quelques jours, les événements vous ont ramenés à la réalité. La semaine dernière, le Gouvernement a ainsi indiqué, par la voix du Premier ministre, qu'il reviendrait sur la fiscalité de l'énergie, et le Président de la République a annoncé cette semaine qu'il reviendrait sur la question de la CSG des retraités.

sur le renforcement de la justice fiscale. Ces mesures s'ajoutent, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, à l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant que le Premier ministre a annoncée la semaine dernière. Mardi dernier, le Sénat a bien voulu accepter la seconde délibération demandée par le Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2019, afin de permettre l'accélération de la hausse de la prime d'activité.

aux assemblées de se saisir très rapidement, dans le calendrier contraint qui est le nôtre, d'un texte reprenant les promesses qui ont été faites devant les Français, tout en tenant compte des exigences constitutionnelles et des conditions de travail de la représentation nationale. Comme vient de l'indiquer le Premier ministre, un projet de loi sera examiné

Monsieur le ministre de l'agriculture, vous connaissez, je le sais, la détresse extrême de nombreux agriculteurs, qui souffrent d'un revenu beaucoup trop faible. Voilà dix-huit mois,

si nous laissions se dérouler les négociations commerciales telles qu'elles se passent depuis dix ans, nous allions dans le mur : 340 000 agriculteurs, 16 000 entreprises de transformation, 4 centrales d'achat ! Ce constat, nous le partageons toutes et tous. Après les

du budget 2019. Je vous l'ai déjà dit ici, c'est une réalité. Les chiffres sont têtus, le budget est têtu, et le rapporteur général du budget ne me démentira pas. Ensuite, nous voulons aller beaucoup plus loin, et pour aller beaucoup plus loin, monsieur Raison, nous avons besoin de tous. Comme sénateurs de la majorité, vous aimez les agriculteurs ; vous en étiez un. Vous voulez que les choses réussissent. Alors, monsieur Raison, aidez-nous à faire en sorte qu'elles réussissent ; aidez-nous à convaincre l'ensemble des acteurs de la chaîne

Vous n'avez rien touché aux charges. Il y a des années que le gazole est détaxé, parce qu'on ne brûle pas le gazole sur les routes. Monsieur le ministre, empoignez deux sujets prioritairement les charges des agriculteurs, auxquelles j'associe la complexité administrative, mais n'oubliez pas la réforme de la politique agricole commune, qui procure une partie des recettes des agriculteurs. Le prix n'est pas le levier du politique ; le levier du politique, ce sont les charges et la politique agricole commune.

crise migratoire historique qu'elle traverse, de nouvelles interrogations émergent. À force d'inaction, parfois même de déni de réalité, la question migratoire n'a pas été gérée, comme nous l'ont d'ailleurs rappelé les oubliés de la croissance, les perdants de la mondialisation. Dans ce contexte particulièrement tendu, de nombreux Français découvrent le Pacte global pour les migrations sûres, ordonnées et régulières porté par l'ONU. Si pays d'accueil, pays de transit et pays d'origine peuvent au moins s'accorder sur l'intitulé du pacte, il reste que le contenu et la méthode ne laissent pas d'interroger, voire d'inquiéter, car le texte sur lequel s'engage notre pays n'a rien d'anodin. Les signataires y prennent l'engagement de réaliser 23 objectifs, déclinés en près de 200 mesures spécifiques, dont la mise en oeuvre sera, en outre, surveillée par un mécanisme de suivi et d'examen. Comme souvent, les inquiétudes sont balayées, voire méprisées par les tenants du pacte, qui présentent les esprits sceptiques comme, au mieux, mal renseignés ou, au pire, mal intentionnés. De surcroît, le plus élémentaire des réflexes démocratiques aurait dû être, pour le Gouvernement, d'informer la représentation nationale de ce projet et d'en débattre avec elle avant de prendre définitivement position. Dès lors, monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement a-t-il conscience qu'en procédant de la sorte il contribue à un affaiblissement démocratique renforçant le sentiment que les peuples n'ont plus leur destin en main

C'est un document dont le préambule réaffirme la souveraineté des États pour établir leur politique migratoire, et qui vise à rappeler la coresponsabilité entre les États de transit, les États d'origine et les États de destination. Ce document, qui, d'ailleurs, a un caractère non contraignant- c'est écrit noir sur blanc, et cela a été rappelé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres -, a comme vertu d'être une boîte à outils, dont les États peuvent s'emparer pour faire face à ce défi mondial. Ce défi, on ne peut pas le résoudre tout seul. Le Gouvernement a pris soin, naturellement, d'informer le Parlement. J'ai d'ailleurs entre mes mains le texte qui a été transmis au Sénat,

une résolution européenne du Sénat sur le suivi des conclusions de la commission d'enquête sur Schengen- M. Reichardt a beaucoup travaillé sur le sujet -rappelait un certain nombre de principes, invitant le Gouvernement à s'y tenir. Sont notamment mises en avant « la coopération approfondie et fructueuse avec les pays d'origine »- c'est un des fondements du pacte -, et la « nécessité de négocier avec les pays tiers sur le retour et l'admission »- cela tombe bien aussi, c'est l'objectif 21 du pacte ! C'est donc fort de votre inspiration que le Gouvernement s'est rendu à Marrakech pour approuver ce pacte pour la réplique. Merci, monsieur le secrétaire d'État, de cette réponse, mais je crois quand même que, dans le contexte particulièrement tendu que nous traversons, et les dernières semaines viennent de nous le confirmer, les Français en ont assez de la verticalité comme mode de gouvernance. Ils veulent plus d'informations, de démocratie, de démocratie, et un État qui prenne ses responsabilités. Il faut conclure. Dès lors, je crois qu'il n'appartient pas à des experts de se substituer aux élus nationaux et de préparer, en sous-main,